Il impose à ces organismes de veiller au respect de ces principes par les personnes qui participent à l'exécution du service public. J'y insiste : « veiller ». D'après le, c'est un verbe qui définit un état dans lequel nous ne sommes pas endormis. C'est une bonne chose.

principes dans le cadre de son pouvoir disciplinaire à l'égard des agents qui sont sous sa responsabilité, afin, tout simplement, de passer d'un état passif à une attention bienveillante.

respecter les obligations qui incombent à ses salariés. Cela comprend évidemment les mesures disciplinaires. Cette mention permet en outre à l'employeur de procéder par d'autres voies, en adaptant les stipulations du contrat de travail, par exemple. Une partie de ces amendements est ainsi

Sur un sujet aussi sensible et fondamental, notre législation doit être claire et ne pas laisser la place à des ambiguïtés ou à des sous-entendus. La marge interprétative doit être très limitée. Or, de ce point de vue, la rédaction actuelle de l'article 1 du projet demeure insatisfaisante en raison de l'ajout de l'adverbe « notamment ». Il ne s'agit pas d'un point de détail simplement rédactionnel : l'introduction de ce mot risque de donner lieu à une lecture qui étendra la portée de ces dispositions au-delà des opinions politiques et religieuses. religieuses. Pourquoi ne pas viser strictement la manifestation d'opinions religieuses ou politiques, le respect de la liberté de conscience et le traitement égal et digne des usagers ? L'ouverture que suggère ce « notamment »

Il nous semble important de garder un parallélisme entre ces deux dispositions pour bien faire comprendre qu'elles renvoient aux mêmes obligations à la fois pour les fonctionnaires et pour les salariés des entreprises auxquelles a été confiée une délégation de service public.

de la laïcité, et je pense qu'il serait très utile aujourd'hui de retrouver cette même volonté de défendre la République et la laïcité. Vous citez Jules Ferry, mon cher collègue ; permettez-moi de citer Ferdinand Buisson, en 1911, Buisson, en 1911, dans son : « Dans l'évolution de la démocratie, les instituteurs de demain continueront à peu près le même office qu'avaient rempli ceux d'hier à l'égard de la République naissante. Ceux-là avaient frayé la voie aux réformes politiques ; ceux-ci l'ouvriront aux réformes sociales. »

Si elle était maintenue, nous aurions dans notre droit des rédactions divergentes entre, d'une part, l'article 25 de la loi de 1983 relative à la fonction publique, qui impose aux fonctionnaires de s'abstenir, dans l'exercice de leurs fonctions, de manifester leurs opinions religieuses, d'autre part, qui impose aux salariés participant à une mission de service public de s'abstenir de manifester leurs opinions politiques et religieuses. Rien ne justifie cette différence de rédaction, alors même que l'objet de ces deux articles est le même. Lors de l'examen en commission des lois, Mme la rapporteure s'était montrée sensible à cette nécessité de faire converger les deux rédactions, deux rédactions, et la commission avait d'ailleurs adopté un de nos amendements, identique à un amendement déposé par Alain Richard, pour mentionner à l'article 1 l'exigence de traiter de façon égale toutes les personnes et de respecter leur liberté de conscience et leur dignité, obligation qui s'impose déjà aux fonctionnaires en vertu de la loi de 1983. Avec cet amendement, nous proposons d'aller au bout de cette logique uniformisant les rédactions de ce projet de loi et de la loi de 1983. Un objectif qui nous paraît d'autant plus facile à atteindre que la mention des opinions politiques n'est pas utile, puisqu'elle est déjà couverte par l'obligation de neutralité. De plus, elle peut prêter à confusion.

chacun respecte une obligation de neutralité, qu'elle soit religieuse, politique ou philosophique. Sur l'amendement de Roger Karoutchi, c'est vrai, nous sommes

à l'université. Ce texte ne dit pas exactement s'il s'applique à tous les fonctionnaires et, en tant que professeure d'université, j'aimerais bien quelques explications sur ces trois amendements.

la terminologie qu'il emploie s'éloignerait trop des textes précédents, et notamment de la loi de 1983, tandis que nous-mêmes souhaitons que le texte soit identique pour éviter toute confusion. Cette remarque justifie que nous maintenions notre amendement.

parce que j'ai du mal à imaginer que l'on puisse obliger à un enseignement religieux et ne pas permettre, dans le même temps, de manifester des opinions religieuses, philosophiques et politiques. Cela va être un petit peu compliqué. À mon sens, dans tout le texte, dans tous les amendements qui vont suivre, il faudra, chaque fois, se poser la question de l'application à l'Alsace-Moselle, où il y a un régime particulier. Si l'on ne dit pas que ce que nous votons ne s'applique pas à l'Alsace-Moselle, cela va s'y appliquer. La parole est

certains signes et vêtements sont parfois instrumentalisés, en dehors de toute connotation religieuse, en vue de marquer des discriminations sexuelles, et notamment dans le but d'inférioriser les femmes.

au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations définit de manière claire et détaillée ce qu'est une discrimination. Elle érige ce principe en l'un des fondements les plus élémentaires de notre droit et de notre société. Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 1 du projet de loi précise bien que toutes les personnes doivent être traitées de façon égale dans le cadre du service public. Néanmoins, il paraît nécessaire d'aller au-delà, en précisant que tout traitement doit être fait sans discrimination. Nous avons ici l'occasion de réaffirmer un principe qui est au coeur de notre pacte républicain. L'objet de ce projet de loi étant précisément de conforter le respect des principes de la République, il est indispensable que celui de la non-discrimination y soit inscrit.

a été consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Si l'article 1 du projet de loi vient réglementer l'exercice du service public, notamment du point de vue des manifestations d'opinion, il est nécessaire que l'indépendance universitaire soit préservée. Aussi, nous souhaitons préciser que les dispositions de l'article 1 ne doivent pas faire obstacle au respect du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.

principalement applicables aux salariés de droit privé. Les agents publics, catégorie à laquelle appartiennent les enseignants-chercheurs, demeurent soumis aux obligations déjà prévues par les statuts de la fonction publique.

proposons d'aller un petit peu plus loin et d'inscrire dans la loi qu'un organisme qui entre aujourd'hui dans le périmètre de l'article 1 resterait soumis au respect des principes de laïcité et de neutralité quand bien même il n'y entrerait éventuellement plus, parce que son régime juridique aurait évolué. Pour le dire autrement, il s'agit de poser le principe selon lequel le passage d'un organisme du service public vers le domaine concurrentiel est sans conséquence sur l'application du principe de laïcité à cet organisme. Il s'agit en quelque sorte d'un mécanisme de cliquet, qui vise à garantir que le passage du service public au champ concurrentiel ne sera pas l'occasion d'une baisse d'ambition en matière de respect du principe de laïcité.

en application du présent article. Dans l'autre hypothèse, s'ils ne devaient plus être chargés de l'exécution d'un service public, il ne serait pas normal de les traiter différemment des autres entreprises. Dès

ouvert au public séparés pour les hommes et les femmes. Il s'agit en particulier de créer une police spéciale du maire pour la répression des discriminations à l'accès des établissements publics accueillant du public. En vertu de cette police spéciale, serait d'abord tenu d'informer le contrevenant des sanctions encourues. Cette obligation, inspirée de ce qui existe en cas de constat d'infraction en matière de déchets, donnerait en outre un argument aux maires sollicités par des associations qui réclament, sans aucune justification réelle, la mise à disposition de piscines publiques dans une intention discriminatoire. Le maire pourrait aussi, dans le respect des droits de la défense, prononcer des sanctions administratives, bien entendu sans préjudice de ce que pourrait décider la justice, saisie parallèlement fermeture de l'établissement public ou astreinte journalière. Au passage, il est précisé dans cet amendement qu'il y a discrimination en cas d'accès autorisé selon des horaires particuliers. Serait ainsi levée toute ambiguïté éventuelle sur le fait qu'il s'agit là d'une discrimination.

Je voudrais donc simplement expliquer pourquoi j'ai souhaité le présenter. L'objet de l'article 1 de ce texte est bien entendu de garantir la neutralité des services publics, quel qu'en soit le mode de gestion.

Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.

Ainsi, rien n'interdit le port de signes religieux. Je tiens à souligner que je parle ici de tout signe religieux ! Aux termes de cet amendement, les règlements de ces établissements devront garantir le respect de ces principes de neutralité et de

d'autres peuvent céder à des tentations clientélistes, voire promouvoir une vision de la société contraire à nos principes républicains. Je veux en prendre un exemple. Ces dernières années, dans mon département, la ville de Grenoble, comme d'autres villes ailleurs en France, a été le théâtre d'actes de désobéissance civile de la part de militantes en burkini qui ont enfreint les règlements intérieurs des piscines au nom de la liberté des femmes à vivre leur foi comme elles l'entendaient. Ces actes de provocation médiatisés ont créé une vive polémique nationale. Le maire écologiste de Grenoble n'est jamais sorti de son ambiguïté et il en a appelé à la responsabilité de l'État, déclarant : « Si c'est une question de laïcité, le Gouvernement doit prendre position. »

ailleurs, monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez déclaré que, sous couvert de combattre l'islamophobie, certaines associations font pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir des règles compatibles avec la charia. Nous le savons tous, cette pression est de plus en plus forte en France ; il est de la responsabilité de l'État de ne pas laisser les maires seuls en première ligne. De petites compromissions en grands renoncements, le risque est de voir les digues progressivement céder au gré des spécificités sociologiques et politiques des territoires.

par principe, comme vous le proposez dans cet amendement, de l'expression d'une opinion religieuse. La neutralité ne s'impose pas aux usagers du service public

Au contraire, nous voulons encourager les élus de la République à prendre des dispositions qui sont déjà prévues par la loi, mais qui demandent un peu de courage politique. Je voudrais rappeler, monsieur le sénateur, qu'on n'est jamais obligé de céder au communautarisme et au clientélisme religieux.

dans des conditions pouvant susciter un certain questionnement. Sur le fond, cet amendement pose de nouveau la question de ce qu'est un signe religieux.

Dès lors, le port du burkini par des femmes fréquentant un espace public tel qu'une piscine municipale, s'il constitue effectivement une manifestation religieuse, ne peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue. Je crois que c'est important de s'y tenir.

un signal religieux, mais le signe d'une contre-société sexiste, qui dit aux femmes qu'elles sont inférieures aux hommes et qu'elles doivent se soumettre, et qui veut séparer une communauté des croyants de la communauté des citoyens, de la communauté nationale.

Sur le fond, je serai très bref. La liberté d'expression et la liberté religieuse ne souffrent aucune exception, sauf le trouble à l'ordre public.

peut-être louable et compréhensible à titre individuel, nous interdirions de manière très arbitraire, en tant que législateurs, la liberté d'expression et la liberté religieuse.

l'on divise le monde entre les pudiques et les impudiques. Ce n'est pas possible ! La pression qui est exercée sur les femmes est insupportable, et c'est à nous de les défendre. Puisque nous parlons du principe d'égalité, je citerai l'un de nos collègues qui nous a précédés sur les bancs du Parlement, Henri-Dominique Lacordaire : il disait qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime- c'est le cas aujourd'hui -et la loi qui protège. Pour protéger l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut voter l'amendement de Michel Savin

On peut croire en une religion, ne pas croire, ou être agnostique. Mais réduire, dans tous nos discours, le fait religieux et les croyances religieuses à des considérations textiles, cela n'a aucun sens

nous n'arrivons pas, et vous n'arrivez pas, à en capturer la réalité. On prend des mesures générales qui auront des conséquences sur toutes et sur tous, alors qu'elles ne visent qu'une minorité : c'est le contraire de la loi

des règles particulières devaient être prévues pour les accompagnants de sorties scolaires parce qu'ils étaient des agents bénévoles du service public. Vous nous avez démontré

qu'en ce qui concerne notre groupe communiste républicain citoyen et écologiste, mais j'imagine aussi pour nos collègues de gauche, nous aimons la République autant que vous ! Que la chose soit dite !

Un projet totalitaire a besoin de symboles. Il ne faut pas être naïf : nous avons bien là un symbole totalement contraire à la République,

que, dans la suite du débat, vous trouverez des exceptions pour que ce principe universel ne s'applique pas, notamment quand il sera question d'enseignement.

Premièrement, le texte dont nous débattons ce soir, monsieur le ministre, concerne bien le respect des principes de la République.

je ne voulais pas me focaliser sur une religion.. Quand j'ai travaillé sur ce texte, j'ai discuté avec de jeunes femmes de confession musulmane

qui, comme je l'ai dit précédemment, assure la neutralité des pouvoirs publics à l'égard du culte et un traitement égal aux diverses expressions Cet amendement vise à rappeler que la République, qui garantit la liberté de conscience, reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester sa conviction religieuse en public, tant que l'ordre public est préservé. en même temps à réaffirmer la garantie de la stricte neutralité des personnes exerçant une mission de service public à l'égard des usagers, quelles que soient leurs convictions religieuses. Enfin, n'oublions pas que, parfois, le séparatisme ne naît pas d'une volonté d'opposition aux principes de la République. En revanche, les pouvoirs publics, par leur désengagement dans certains territoires, par le manque de financement des services publics et par le manque de considération accordée aux difficultés de nombreux Français, créent d'eux-mêmes ce séparatisme. Il convient donc de réaffirmer qu'il revient à tout organisme de droit public ou privé chargé de l'exécution d'un service public de garantir la mise en oeuvre effective des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité, de laïcité et de mixité sociale dans l'exercice de ses compétences. L'amendement

Pour des raisons sociales, politiques et religieuses, les femmes se couvrent de gré ou de force la tête et une partie du visage. Elles marquent ainsi un terrible aveu : celui de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Cette conception contraire à tous nos principes et même à notre devise républicaine pourrait rester personnelle si elle n'était pas devenue un enjeu politique depuis une quarantaine d'années. Voiles au lycée, à l'université, au travail, dans la rue, etc. Voile, hidjab, burqa, niqab, burkini : tant de mots et tant de débats qui n'auraient jamais dû se tenir en France. Peut-être que le jour où nous ne débattrons plus du voile nous pourrons réfléchir aux moyens de financer la recherche en vue de la création d'un vaccin contre un virus qui nous pourrit la vie. C'est ce que je vous propose dans cet amendement : interdire le voile dans l'espace public et mettre fin à tous ces débats. Ainsi, la règle sera claire. Le voile doit être interdit dans l'espace public parce que, outre son caractère discriminant, il sert aujourd'hui d'étendard aux revendications communautaires et islamistes.

Il n'y a qu'une seule loi en France, celle de la République, et qu'une communauté, la communauté nationale. Pour les islamistes, le voile constitue aussi un moyen de pression exercé sur celles qui ne le porteraient pas : elles sont marginalisées, moquées, parfois insultées et frappées parce qu'elles refusent de se soumettre. le voile serait un rempart contre la violence : plus d'une musulmane sur quatre le porte pour se sentir en sécurité. Il s'agit non plus de séparatisme, mais d'une véritable domination domination exercée par les islamistes. Ceux-ci ne veulent pas vivre en dehors de la République, ils veulent que la charia supplante nos lois, en commençant par l'asservissement des femmes. Les élus que nous sommes ne peuvent pas cautionner cette situation. Nous devons tendre la main à toutes celles qui ne rêvent que d'une chose : être libérées et s'affranchir du voile. C'est pour libérer toutes les incarcérées dans une geôle de textile- une étoffe peut tout aussi bien priver de liberté que des barreaux -et éradiquer toute marque de conquête islamiste que nous devons, mes chers collègues, agir en votant cet amendement.

L'interdiction pour les mineurs de porter dans l'espace public tout signe religieux ostensible aurait pu constituer un signal fort envoyé à notre jeunesse. Celle-ci aurait pu y voir une garantie de la préservation de son insouciance et de sa liberté. Dans quelle mesure une République laïque peut-elle tolérer que des enfants manifestent des signes religieux au su et au vu de tous ? Ce n'est pas aux parents d'imposer des dogmes aux enfants. Aussi, il est essentiel qu'existent des espaces protecteurs, vecteurs d'émancipation, Le présent amendement vise à interdire, dans l'espace public, le port par des mineurs de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Dans cette perspective, il est indispensable d'empêcher tout moyen d'inférioriser l'enfant, notamment la jeune fille, au travers d'un vêtement qu'on lui impose.

conformément à la convention de l'Organisation des Nations unies relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a trente ans. Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes au regard sexualisé des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ? Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge ou de jeunes n'ayant pas atteint l'âge du consentement ? Le voilement des mineurs peut représenter des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.

Alors quand elle croise aujourd'hui une femme qui le porte, elle dit que cela lui est insoutenable. Voici ce qu'elle écrit : « Le voile est un symbole qui ôte toute capacité à la femme d'être un être pensant. Quand un seul de ses cheveux peut susciter le désir sexuel le plus fruste de l'homme, elle est réduite à un appât sexuel. Ce symbole pornographique autorise toute forme de violence à l'encontre des femmes et les place dans le non-droit. Quand on voile une petite fille, on lui inculque la culpabilité de sa sexualité féminine, on lui dit que ses cheveux et les formes de son corps peuvent à tout moment faire perdre le contrôle de soi aux hommes. Je demande qu'au moins dans les pays démocratiques, le port du voile par des mineures soit sanctionné. Cela relève des droits de l'homme et de la protection des mineurs. » J'ajoute que cet

la France est une République laïque " [ ...] interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». Aussi, j'ai rectifié mon amendement

: La parole est à M. Bernard Fialaire. Le présent amendement vise à interdire, dans les services publics, le port des signes ou de tenues par lesquels les mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

à ces jeunes filles et même à toutes ces femmes qui, à travers le monde, risquent avec courage leur vie en refusant de porter un voile, afin de sentir le vent dans leurs cheveux. C'est le moment de le faire, mes chers collègues ! Nous n'allons pas encore attendre je ne sais quel texte.

En cinq ans, les demandes adressées au Défenseur des droits ont bondi de plus de 40 % ; on y retrouve, pêle-mêle, des constats de non-accès au service à cause d'une dématérialisation à marche forcée, des fractures fortes entre territoires, dont les services publics disparaissent petit à petit, mais aussi des difficultés de plus en plus grandes

sécuritaire. Le responsable allemand qu'il était avait compris que le recul des politiques publiques engendre une crise de confiance vis-à-vis de l'État, puis la défiance et, pour finir, le rejet de celui-ci. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que les troubles sociaux se déclenchent généralement dans les territoires abandonnés

prêteront serment solennellement pour certifier de leur adhésion à la République et à ses principes. Une telle disposition est bienvenue, mais elle suggère automatiquement une interrogation pourquoi se limiter à cette liste restreinte de fonctionnaires ? Pourquoi ne pas étendre cette disposition ? Tous les fonctionnaires doivent être sensibilisés aux principes les plus essentiels de notre République, tels que ceux qui sont affirmés dès l'article 1 de la Constitution, selon lequel « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale[, qui] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion [et] respecte toutes les croyances

Ce serment républicain sera par conséquent étendu à tous les agents de la fonction publique qui auront, tout au long de leur carrière, à se soumettre aux obligations de neutralité du service public.

qui figure actuellement dans la prestation de serment du personnel de l'administration pénitentiaire, nous paraît importante, car elle met l'accent sur le fait que les principes de la République, auxquels il sera prêté serment, ne sont pas désincarnés ; ils doivent se traduire dans la réalité du quotidien des Français. Tel est le sens de cet amendement.

que les conseillers soient conscients, dès leur prise de fonction, de leur responsabilité dans la représentation locale de notre démocratie républicaine, qui est laïque et séparée des cultes depuis 1905. Ainsi, cet amendement tend à instituer un serment républicain que prononceraient les conseillers municipaux nouvellement élus.

Requier. Le code de la sécurité intérieure permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l'embauche ou les décisions d'affectation de leurs salariés « d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure est essentielle, car elle permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n'est pas en cours de radicalisation religieuse. Toutefois, en cas d'avis négatif, l'employeur est dans l'obligation de proposer un reclassement à l'employé